La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire. Dans la discussion du texte de la commission,

un détour par la question des opérateurs alternatifs avant un retour d'expérience. Il est tout de même temps, en effet, de se libérer quelque peu des illusions de l'ouverture à la concurrence. à la concurrence. Dans le champ du ferroviaire ouvert à la concurrence, il se passe ce qui a pu se passer dans d'autres services publics ayant subi le même traitement. On pense aux renseignements téléphoniques, à l'oligopole cartellisé de la téléphonie mobile ou au réseau de bus promus par la loi Macron. Nous nous retrouvons très vite avec une situation déjà connue : en lieu et place d'un monopole public animé par les vertus et qualités du service public, nous avons un oligopole d'entreprises. Cet oligopole de structures, de masse critique évidente, directement en lien avec des opérateurs ferroviaires venus de l'étranger- la SNCF, quant à elle, travaille au Royaume-Uni ou encore en Allemagne -, n'a rien à voir avec une logique de PME. de PME. Il s'arrange sur les prix, le partage du marché et les conditions de service offertes à la clientèle. Examinons, par exemple, le cas de la téléphonie mobile. Nous avons quatre opérateurs : Orange, l'opérateur historique dans notre pays, dont le capital, fruit des efforts de l'ensemble de la Nation, a été dilapidé, Free, SFR et Bouygues Telecom. Ce dernier opérateur est, certes, une société spécialisée, mais ses liens avec un groupe multifonctions en font, en quelque sorte, la poule aux oeufs d'or destinée à en permettre la rentabilité. Les opérateurs de la téléphonie mobile se sont accordés sur un, évidemment évidemment dissimulé au grand public, lorsqu'il fallut assurer la montée en puissance du marché du téléphone mobile et équiper à peu près tout habitant de ce pays âgé d'au moins douze ans d'un appareil de cette nature. Maintenant que nous sommes parvenus à la quasi-saturation du marché en termes de nombre d'abonnés, la concurrence se détermine sur les variables sociales et la dégradation continue des conditions de travail des salariés du secteur. Le téléphone mobile, quand il est, va de pair avec le en matière de critères sociaux. Pour autant, cette concurrence organisée et structurée n'a pas répondu aux attentes de ceux qui ont ouvert le secteur à la concurrence en 1996, à savoir garantir une égalité d'accès aux services de téléphonie mobile, avec tout ce que cela implique pour la vie quotidienne. La parole est à Mme Angèle

Lors des débats devant l'opinion publique, le Gouvernement, par votre voix, madame la ministre chargée des transports, s'était engagé à ne pas passer par le biais des ordonnances sur la question de l'ouverture à la concurrence du marché des transports ferroviaires de voyageurs. Il reconnaissait ainsi la nécessité du rôle du Parlement sur ce sujet. Si le Gouvernement souhaite assurer la cohérence de ses déclarations, il ne peut pas conserver en l'état l'article 3, qui tend à lui accorder autorisation de rédiger des ordonnances pour gérer l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Quel est l'avis de la commission ?

Cette fois, l'affaire est diablement sérieuse. Il s'agit de créer les conditions de transfert intégral des équipements, des femmes et des hommes du rail au bénéfice des sociétés parcellisant les activités actuelles de la SNCF. est de créer les conditions d'une large ouverture à la concurrence, y compris en procédant à la cession au privé des matériels et personnels de l'actuelle SNCF. Cette logique est en ligne avec une partie de l'organisation interne de la société nationale, dans laquelle les cheminots se trouvent de plus en plus cantonnés sur un réseau donné, par exemple le réseau sud-est ou le réseau nord, sans parler de la spécialisation des trains de banlieue. Ce mouvement vers la spécialisation est nuisible à la cohérence du métier lui-même.

Le règlement européen, comme l'article, n'exclut nullement que l'on procède à une sorte de vente par appartement, permettant d'ailleurs, du point de vue de l'État- je pense notamment aux comptes publics -, qu'une partie de la dette d'investissement portant sur les matériels puisse être gagée sur l'indemnisation de leur cession. Cette dilapidation des actifs du groupe public est une mauvaise manière faite aux usagers, et ce d'autant plus qu'elle risque fort de conduire à l'extrême usure, après l'extrême usage des matériels ainsi transférés. outre, elle s'appuie sur un évident moins-disant social, ouvrant la possibilité, dans le cadre des sociétés ferroviaires banalisées, d'un recrutement de personnels précaires, aux fins de limiter les coûts.

Afin de prendre en compte au mieux les enjeux sociaux, humains et environnementaux de la mise en concurrence d'opérateurs pour l'attribution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, il est nécessaire que l'autorité organisatrice mette en place un processus de concertation, de dialogue social et de négociation impliquant les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel des entreprises exploitantes existantes. Ce processus inclut notamment une consultation préalable à la rédaction du cahier des charges de l'appel d'offres, puis, après l'attribution du marché, dans la période précédant le début de l'exploitation par l'opérateur choisi. La concertation et le dialogue social auront notamment pour objectif de corédiger un « plan de développement humain concerté », qui sera annexé au cahier des charges de l'appel d'offres et fera l'objet d'un suivi régulier sur la durée du contrat de service public. Ce plan comportera, en particulier, des dispositions permettant de s'assurer de la loyauté des pratiques sociales de l'opérateur et de leur conformité avec les engagements pris. de définir des clauses sociales et environnementales à inclure dans l'appel d'offres, puis d'en assurer le contrôle et le suivi. La pratique de clauses sociales existe dans les marchés publics dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et s'applique dans le transport urbain et interurbain de voyageurs. L'analyse des effets de ces dispositions montre que, lorsqu'un dialogue intervient entre l'autorité organisatrice de mobilités et les représentants syndicaux, et que ces derniers sont informés en amont des projets de l'autorité organisatrice de mobilités, une concertation et certaines formes de négociation sur l'intégration de clauses sociales dans les spécifications des marchés permettent de trouver des solutions à d'éventuelles difficultés et d'anticiper les effets sociaux d'un possible changement d'opérateur. Prévoir que les spécifications des marchés incluront des clauses sociales et que celles-ci feront l'objet d'une négociation permettra d'anticiper les difficultés liées aux transferts éventuels des marchés et des salariés à un nouvel opérateur, ainsi que de faciliter un transfert se réalisant dans de bonnes conditions humaines et sociales, donc de manière favorable en termes d'objectifs de service au public. Quel est l'avis de la commission ?

qu'un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices et des représentants des organisations syndicales- c'est un gage de concertation -, précisera les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les marchés

sens. Il s'agit de supprimer le renvoi par cet article à une énième ordonnance des conséquences du refus par un salarié de son transfert vers un opérateur concurrent. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément central de la réforme ferroviaire, qui mérite d'être traité. Comme nos débats vont encore durer quelques heures, je prends un peu d'avance, madame la ministre

Il en est ainsi de l'alinéa 6, qui permet le recours aux ordonnances pour déterminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par la SNCF pour l'exécution d'un contrat de service public ferroviaire attribué avant 2023. Il s'agit notamment du matériel roulant et des ateliers de maintenance. Que l'on parle du matériel reçu, c'est une chose, mais évoquer le matériel créé ou acquis par la SNCF semble bien trop large. Cette question est trop importante pour être renvoyée à plus tard, d'autant qu'elle est déjà traitée dans le nouvel article 2 . Nous ne Nous ne pouvons accepter le recours à une ordonnance sur un sujet aussi structurant pour l'avenir de SNCF Mobilités, qui se verrait ainsi dépouillée de ses biens en même temps que de ses contrats. les régions ont largement participé au financement des matériels roulants, mais est-ce une raison suffisante ? Pourquoi ne pas laisser les nouveaux entrants réaliser des investissements ? Pourquoi leur permettre de récupérer les matériels, les agents, les ateliers ? Quelle sera donc la différence si tout change dans une stricte continuité ? Par ailleurs, une telle disposition n'est pas sans poser des problèmes pratiques. En effet, les ateliers de maintenance servent souvent à de multiples tâches, et pas exclusivement aux transports régionaux. Il semble dès lors qu'il soit compliqué de prévoir leur reprise par les régions sans créer de difficultés pour l'organisation de SNCF Mobilités. Reste enfin une question essentielle, celle du matériel amianté. sujet l'attention de l'ensemble du Sénat. Les régions risquent d'hériter de charges qui vont se révéler des cadeaux empoisonnés, si je puis me permettre cette expression, à l'image du matériel lorsque celui-ci est obsolète. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons légiférer à l'aveugle sur ces questions, même si le champ de l'habilitation a été précisé en commission. Pour cette raison, nous proposons la suppression de cette habilitation. C'est un sujet très sérieux

insiste, les régions doivent être en mesure de récupérer le matériel roulant avec le carnet d'entretien à jour et les plans de maintenance actualisés. La reprise du matériel roulant nécessite nécessite un transfert du plan de maintenance, de l'historique de la maintenance et des consommations d'énergie, de la liste des pièces de rechange et des pièces de parc mises à disposition, ainsi qu'un état des lieux contradictoire avec l'exploitant sortant. L'amendement

des autres biens utilisés par SNCF Mobilités dans le cadre des services conventionnés. Nous savons que l'acquisition des matériels roulants et l'accès aux ateliers de maintenance pourraient constituer des barrières à l'arrivée de nouveaux opérateurs.

la commission a déjà précisé que le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance devait s'accompagner du transfert des éléments nécessaires à l'exploitation de ces biens, à l'appréciation de leur état et de leur valeur, dont les carnets d'entretien à jour. Cet amendement vise à ajouter la transmission du « retour d'expérience La rédaction de la commission est déjà assez complète, et je ne vois pas très bien à quel document précis font référence les termes « retour d'expérience ».

n° 122 rectifié vise à inclure les plans de maintenance dans les éléments nécessaires à l'exploitation des biens transmis. Il s'agit d'une question complexe, vous le savez, monsieur Longeot, car il faut trouver un équilibre entre la nécessité de fournir les informations indispensables et la protection du secret industriel et commercial. Nous en avons déjà parlé. Ce sujet mérite donc, à mon sens, des concertations entre les acteurs directement concernés. De notre côté, nous n'avons pu

-aux carnets d'entretien, sans préjuger de ce qui pourra être décidé par la suite, car l'ordonnance pourra très bien prévoir la transmission de ces plans de maintenance même si nous ne le précisons pas ici. Par ailleurs, la notion même de plan de maintenance me semble devoir être définie.

Madame Assassi, vous avez mentionné la question des matériels amiantés.

en train de parler sont des dispositions techniques ou de mise en oeuvre. Les principes, eux, ont été clairement inscrits dans le texte. Il me paraît logique de laisser

des savoir-faire industriels, qui sont le résultat des années d'expérience de la SNCF dans ce domaine et n'ont pas à être transférés aux concurrents. La rédaction actuelle précise largement les choses.

L'autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu'elle ne reprend pas à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées.

conventionner avec un opérateur de services librement organisés pour assurer une continuité de parcours sur leur territoire, afin, par exemple, d'assurer des dessertes TGV au-delà des seules métropoles, de desservir ainsi finement le territoire. L'habilitation à légiférer par ordonnance a pour objet de préciser les règles applicables dans ce cas. Il s'agit par exemple d'exclure la possibilité que les matériels roulants soient transférés vers l'autorité organisatrice, ce que la

de cet amendement aurait pour conséquence d'élargir de façon substantielle le champ de l'habilitation, puisqu'elle permettrait au Gouvernement de déterminer

me semble excessive. J'ai demandé au Gouvernement- je l'ai fait sur l'ensemble des habilitations à procéder par ordonnance -pourquoi il sollicitait une telle habilitation. Depuis le départ, il m'a été répondu qu'il s'agit de traiter la question des biens utilisés dans le cadre de services conventionnés et de services commerciaux.

En l'absence d'éléments d'information complémentaires sur cette demande d'habilitation, et compte tenu du caractère très large de la rédaction proposée, nous ne pouvons accepter cet amendement. La commission a donc émis un avis défavorable

Par ailleurs, il faut bien dire que personne n'est mieux placé que les usagers d'une ligne pour faire remonter les difficultés de circulation, mais aussi des pistes d'amélioration et d'aménagement des horaires ou des quais d'arrivée par exemple- nous avons tous été confrontés à ce ailleurs, ne peut mieux expliciter les limites techniques, financières et managériales que les autorités organisatrices de transport. Enfin, il nous semble important et nécessaire d'évaluer l'accessibilité, donc de permettre une représentation des associations de personnes handicapées.

un souci de transparence et de bonne information. Les comités de ligne, qui ont existé entre 2002 et 2008 avant d'être supprimés en 2010, comprenaient des représentants des régions. Quel est l'avis

Quel est l'avis de la commission ? Les comités de suivi des dessertes visent à associer les représentants des usagers aux choix pris par l'autorité organisatrice dans le domaine des services publics ferroviaires. Il me semble donc tout à fait pertinent d'y inclure les associations représentant des personnes handicapées, afin que la problématique de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite soit bien prise en compte- je suis d'accord La présence d'élus des collectivités territoriales concernées permettra aussi de relayer les attentes des usagers de leur territoire- j'en suis tout à fait d'accord. En revanche, la présence des salariés dans ces instances ne me semble pas correspondre à l'objet

je pense qu'il est en effet très important que les représentants des personnes handicapées soient aussi associés à ces comités de suivi des dessertes. En revanche, pour les mêmes raisons que celles exposées par M. le rapporteur,

des dessertes. L'objet de cet amendement est d'intégrer les représentants des associations de protection de l'environnement

Mme la ministre. Quel est l'avis du Gouvernement ?

que nous sommes ouverts. L'idée n'est pas mauvaise. Il s'agit d'assurer la participation des représentants des associations d'usagers à la gouvernance des services de transports publics réguliers, en créant des comités de suivi des dessertes. Cependant, l'article ne nous paraît pas complet. complet. Il recense tous les motifs de consultation des comités, mais oublie de porter une attention particulière aux performances énergétiques et écologiques en matière de dessertes. En effet, l'impératif écologique lié au développement du ferroviaire ne peut être négligé. Il doit au contraire apparaître comme une priorité politique. C'est ce que nous avons ajouté hier. Nous nous avons ajouté hier. Nous proposons donc d'amender cet article en permettant aux comités de suivi des dessertes de disposer d'un bilan sur l'efficacité énergétique et écologique des choix réalisés en matière de dessertes et de service public des transports. En adoptant cet amendement à l'unanimité, nous serions en cohérence avec ce que nous avons voté hier.

a pour objet de proposer une consultation des comités de dessertes sur la performance énergétique et écologique des choix effectués par les autorités organisatrices. Je n'y suis pas opposé. Un tel enjeu doit être pris en compte dans les choix et peut expliquer certaines décisions prises vis-à-vis des

au même titre que l'opérateur historique. Ces comités doivent associer l'ensemble des parties prenantes, particulièrement la représentation des voyageurs. Ces instances doivent davantage se porter sur les que ne le font les instances régionales de concertation actuelles, inclure les gares des villes moyennes et porter sur la gouvernance des infrastructures, mais également sur la coordination des services, l'articulation des modes et l'intermodalité. Quel est l'avis de la commission ? ? Cet amendement a pour objet la création de comités de pôles d'échanges multimodaux. L'idée est évidemment intéressante, mais elle concerne un champ plus large que les seuls transports ferroviaires. Nous savons que nous aurons bientôt une réflexion globale sur ces questions dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Je préfère que nous attendions ce débat pour légiférer sur le sujet et avoir une position harmonisée, après consultation de l'ensemble des parties prenantes, plutôt que d'introduire des dispositions dans le code pour les modifier dans quelques mois.

Cet amendement important vise à mieux associer les territoires. Nous comptons conférer aux régions, départements, communes et EPCI un droit de regard essentiel sur la gestion des dessertes ferroviaires ou des lignes, en allant plus loin que la simple information ou consultation qui sont actuellement proposées. Les collectivités locales, en particulier les régions et les communes, ainsi que les EPCI, ont la charge de l'aménagement du territoire et des transports. Il est impensable de passer outre leur avis avant de prendre des décisions aussi graves et difficilement réversibles que la fermeture de lignes ou de dessertes ferroviaires. Les usagers sont les destinataires du service d'intérêt national qu'est le transport ferroviaire. Ils en sont dépendants pour leur vie professionnelle et personnelle. Il est donc indispensable qu'une négociation s'effectue sur la question des lignes et des dessertes ferroviaires avec les élus locaux. Nous ne pouvons permettre que des villes ne soient plus desservies au motif de la rentabilité. Cela entraînerait un isolement des populations, un accroissement de la fracture territoriale, avec les conséquences politiques délétères que l'on connaît. Inévitablement, pour compenser cela, il sera mis en place, au mieux, un service de cars, nécessairement plus polluant, pour pallier l'absence de trains. Or nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à rebours des efforts écologiques que nous devons effectuer et auxquels la France s'est engagée. Il nous semble donc nécessaire d'accorder plus de poids aux territoires s'agissant de la gestion des dessertes ferroviaires, tant pour notre responsabilité écologique que pour le respect des citoyens.

la consultation sur la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national et l'information sur la consistance des services librement organisés par une entreprise ferroviaire aux comités de suivi des dessertes, qui permettent l'association des représentants des usagers.

départements et communes, elles touchent aussi la vie quotidienne des usagers. C'est pourquoi, dans un souci de meilleure participation des usagers à la décision publique, une telle modification est proposée. La consultation des représentants des personnels a le double avantage de permettre une information claire de personnels et d'informer les collectivités et usagers d'éléments internes qui permettraient un éclairage industriel et social des créations, suppressions ou modifications.

Cet amendement est motivé par les mêmes préoccupations que celui qui vient d'être présenté. L'article prévoit que les collectivités territoriales concernées en cas de modification d'un service d'intérêt national conventionné sont consultées par l'État. Nous considérons que les fédérations nationales d'associations d'usagers des transports doivent être également consultées par l'État en cas de modification de la consistance d'un service national de transport Je vous remercie,

par M. Jacquin, Mme Préville,

Deuxièmement, nous souhaitons ajouter les EPCI à la liste des structures territoriales et administratives informées par les projets de modification des transports. Il est en effet nécessaire que toute entreprise ferroviaire attributaire d'un service de transport librement organisé informe les collectivités concernées des projets, dès lors que ceux-ci ont été actés, dans un délai fixé à six mois. Ce délai raisonnable est garant d'une meilleure réactivité des collectivités face à la modification d'un service : anticipation sur la mobilité, adaptation des zones périphériques, développement des projets urbains.

L'amendement n° 110 tend à prévoir un avis conforme des collectivités territoriales sur les modifications de dessertes conventionnées par l'État. Nous ne pouvons pas mettre l'État sous la tutelle des collectivités territoriales. La commission émet

C'est l'objet même des comités de suivi des dessertes créés à l'article 3 A. Je considère que cette disposition est pleinement satisfaite sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle disposition législative. vise ensuite l'information des comités de suivi de dessertes sur les modifications des services librement organisés. Dans la mesure où il s'agit de services librement organisés, sans financement public, cette contrainte ne paraît pas pertinente. La commission émet pour objet d'imposer de consulter, avant toute modification d'un service conventionné, les associations d'usagers. C'est, là encore, l'objet même des comités de suivi des dessertes créés à l'article 3 A.

vise à fixer à six mois le délai dans lequel l'État et les collectivités territoriales sont informés de la modification d'une desserte commerciale. Je partage évidemment la préoccupation qu'ils soient informés le plus en amont possible, pour pouvoir réagir et, éventuellement, conclure un contrat de service public. C'est une évidence. la fixation de ce délai relève à mon avis du domaine réglementaire, et je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui quel délai on pourrait raisonnablement demander aux entreprises.

sur les services d'intérêt national est d'ores et déjà satisfaite dans le projet de loi. Et comme les services librement organisés ne dépendent d'aucune autorité organisatrice, il n'est pas possible qu'un comité de dessertes soit consulté.

en cas de suppression ou de modification d'un service d'intérêt national. Le texte prévoit également que l'État, en tant qu'autorité organisatrice, devra créer un comité de dessertes qui comprendra des représentants des usagers et qui sera consulté sur la politique de dessertes. Une telle disposition satisfera la demande des En revanche, il ne m'apparaît pas souhaitable que des salariés travaillant pour une entreprise exécutant un service au travers d'une délégation de service public ou un contrat soient préalablement consultés sur la politique d'offre d'une autorité organisatrice. Le Gouvernement Le présent article prévoit la consultation des collectivités en cas de suppression ou pour une modification d'un service d'intérêt national. Le projet de loi prévoit également que l'État en tant qu'autorité organisatrice devra créer un comité de dessertes

possible sur la modification de la consistance d'un service librement organisé. Cet article prévoit en effet l'information de l'État et des collectivités territoriales concernées en cas de modification de la consistance d'un service librement organisé. Les entreprises ferroviaires ayant l'intention de modifier un tel service doivent préalablement en informer les collectivités Nous souhaitons que les fédérations nationales d'associations d'usagers des transports en soient également informées. Quel amendement est pleinement satisfait par la définition de l'objet des comités de suivi des dessertes, qui seront consultés sur la politique de dessertes et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

dans une logique de complémentarité et d'intermodalité. Je mets aux voix

une procédure préalable à l'arrêt du trafic doit s'imposer aux autorités organisatrices, aux entreprises ferroviaires concernées et à SNCF Réseau, afin d'élaborer et de diffuser, sur la base d'éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants, une analyse du trafic et de l'état de l'infrastructure, l'étude de repreneurs éventuels de l'exploitation, une étude d'impact du report sur l'autocar et les autres modes. SNCF Réseau doit diffuser des informations sur le calendrier de l'arrêt du trafic préalablement à celui-ci. Ce dossier préalable à l'arrêt du trafic doit inclure des éléments d'analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d'autres États membres.

L'objectif de cet amendement est déjà en partie satisfait par les dispositions que nous avons introduites en commission, sur l'initiative de Benoît Huré, pour les services conventionnés par l'État. La procédure proposée ici est extrêmement lourde et mélange les problématiques liées à l'état de l'infrastructure avec le choix de poursuivre l'exploitation de services, qui peuvent être dissociés. Par exemple, si une région décide de supprimer un service parce qu'il y a trop peu d'usagers, on ne voit on ne voit pas pourquoi SNCF Réseau devrait coordonner une étude, sur la base d'éléments recueillis par des experts indépendants, sur l'état de l'infrastructure.

sans une concertation préalable. Et je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités, en particulier aux régions, sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions normatives contraignantes qui n'auraient pas de réelle valeur ajoutée. Par conséquent, le

cet amendement vise à prévenir des fermetures de lignes, de dessertes ou la suppression d'un service régional, comme un guichet, de nature à affecter la qualité des services rendus aux usagers. Encore une fois, le service ferroviaire est essentiel pour la mobilité de tous nos concitoyens. Avec cet amendement, nous souhaitons préserver les réseaux du quotidien, dont les régions ont la charge. Ces derniers sont les plus utilisés pour des raisons professionnelles. Ainsi, si les régions ont la compétence transports, elles ne peuvent pas s'affranchir de l'avis des départements et des EPCI dans la définition d'un réseau de dessertes et de services efficaces. Cela nous semble d'autant plus indispensable depuis la fusion des régions en 2015, leur grande taille ne leur permettant pas toujours d'assurer un service au plus proche des besoins des citoyens. Je prends l'exemple de ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, où la suppression de la ligne Grenoble-Veynes-Gap en zone rurale entraînerait une augmentation importante du temps de transport pour aller à l'université ou au travail. Quand bien même des cars remplaceraient des trains, cela créerait des difficultés pour les personnes à mobilité réduite, les cyclistes- cela a été évoqué tout à l'heure -et les poussettes, c'est-à-dire une dégradation certaine de l'offre de transport. Il nous semble donc indispensable que les acteurs communaux et départementaux, ainsi que les EPCI puissent peser dans la gestion des dessertes, des lignes et des services ferroviaires régionaux.

bonne information et de transparence, il est important que les autres échelons des représentations locales soient associés et, surtout, entendus. À la demande de M. le rapporteur, lors de la réunion de la commission du 23 mai 2018, cet amendement, qui visait à l'origine un avis conforme des départements et des communes, tend à se limiter, dans sa présente version, à un simple avis pouvant éclairer le débat sur une création ou suppression de

? Cet amendement vise à prévoir le recours obligatoire au service interne de sécurité de la SNCF, la SUGE, des entreprises ferroviaires pour assurer les missions de sûreté dans les transports. Actuellement, la loi permet, mais n'impose pas, aux entreprises ferroviaires d'avoir recours à la SUGE, ces entreprises pouvant se doter de leurs propres services de sécurité internes pour assurer ces missions. En commission, nous avons prévu la possibilité pour les autorités organisatrices de contractualiser directement avec la SUGE pour assurer des missions de protection des personnes et des biens dans le cas où une entreprise ferroviaire ne disposerait pas de son propre service de sécurité. Cela garantit que la protection des personnes sera assurée, soit par l'entreprise directement, soit par la SUGE. La commission a donc

de recourir à la SUGE, dès lors qu'elle en fait la demande et dans un cadre régulé par l'ARAFER. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui prévoit prévoit en complément de permettre à une autorité organisatrice de faire appel à la SUGE sans avoir à passer par une procédure de mise en concurrence. C'est un peu la même chose que ce qui avait été décidé en 2014 pour les entreprises ferroviaires, mais transposé aux autorités

Gay, sur l'article. Cet article a été introduit par le rapporteur à l'Assemblée nationale et positivement repris par la commission au Sénat. Il tend à prévoir un rapport- cela arrive, monsieur le rapporteur !-sur les lignes les moins circulées, les fameuses lignes pointées du doigt par le rapport Spinetta, qui a préconisé leur abandon. leur abandon. Ne soyons pas dupes ! Nous sommes face à un numéro de duettistes : d'un côté le rapport Spinetta qui demande l'abandon ; de l'autre le rapporteur M. Djebbari qui souhaite, au travers d'un autre rapport, donner du temps au temps et examiner plus précisément l'état de ces lignes. Au milieu de tout cela, le Gouvernement indique qu'il n'est pas question d'abandonner ces lignes par une décision qui s'imposerait de Paris, mais- je dis bien « mais », car toute la nuance est là -que tout cela sera décidé dans le cadre de discussions avec les régions. Autrement dit, le Gouvernement se déchargera sur les régions de l'avenir de ces petites lignes dans le cadre des contrats de plan État-région ... Belle perspective ! Nous considérons, pour notre part, que toute cette agitation autour des petites lignes témoigne de l'absurdité des réformes que vous préconisez et des lettres de missions des différents rapports qui ont été publiés en début d'année. L'intérêt du service ferroviaire n'est traité que sous l'angle économique et financier. En partant de ce point de vue, il est clair qu'il faut au plus vite se débarrasser de tout ce qui n'est pas rentable et que nous n'avons pas besoin, pour le reste, d'un opérateur public ni d'agents publics.

vous nous demandez de vous croire sur parole. Mais nous avons été échaudés par trop de plans de relance qui n'ont jamais été financés et par les décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de l'État : abandon de l'écotaxe, poursuite des concessions autoroutières, etc. Toute la réforme repose en réalité sur des efforts de productivité demandés à la SNCF, appelés à compenser le sous-financement de l'État pendant quarante ans. C'est impossible, d'autant que vous placez l'entreprise publique en situation de perdre des marchés. Exploiter des lignes non rentables, cela demande des investissements publics, donc un engagement public en faveur du transport ferroviaire. En prônant l'ouverture à la concurrence, au contraire, vous laissez la main au privé sur la satisfaction de besoins d'intérêt général. Nous sommes donc extrêmement inquiets sur l'avenir de ces lignes, qui participent au maillage et au désenclavement des territoires, donc au dynamisme économique des régions. Nous attendons, madame la ministre, des engagements extrêmement forts de votre part sur cette question.

le service pour les usagers et les acteurs économiques que d'apporter une réponse structurante au défi de l'attractivité de l'ensemble des territoires et des bassins de vie, est fondamentale. Elle passe par la réhabilitation des petites lignes ferroviaires aujourd'hui durement affectées par des retards d'investissements chroniques. Malgré la politique mise en place par SNCF Réseau, dans le cadre de son contrat de performance signé avec l'État, afin de réduire le déficit chronique de l'établissement public, qui a confirmé le désengagement du gestionnaire des infrastructures sur les lignes capillaires depuis déjà plusieurs dizaines d'années, l'exigence s'impose à l'État d'engager une réflexion pour assurer la pérennisation de ces lignes sur le temps long, d'identifier dans un rapport dans un rapport remis au Parlement les modes de financement de ces lignes et de mettre les moyens financiers nécessaires pour en assurer la réhabilitation, en particulier avant tout transfert de la propriété de ces lignes aux régions volontaires.

initiale. Nous partageons pleinement les préoccupations de notre collègue Gremillet, auteur de l'amendement, sur la nécessité d'une nouvelle classification

tend effectivement à réécrire totalement l'article en changeant finalement la nature de ce qui est visé. L'article, tel qu'il figure aujourd'hui dans le projet de loi,

que les montants sur la base desquels ces contrats avaient été établis n'étaient pas du tout conformes aux besoins pour la rénovation de ces lignes. Votre proposition me paraît perdre

en vue de la préparation des prochains contrats de plan. De surcroît, je suis gênée par le deuxième alinéa de votre amendement, car il vise un transfert de propriété des lignes aux régions, ce que je ne n'approuve pas. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de prévoir

contribution à l'aménagement du territoire, le tout, en concertation avec les autorités organisatrices. L'objectif est d'aller plus loin que les mesures UIC 7 à 9, qui sont

l'objectif. On passe d'un diagnostic, qui me semble indispensable dans la perspective de la préparation des prochains contrats de plan, à un état des lignes les moins circulées en vue d'établir une classification. La rédaction actuelle

? Cet amendement vise à prendre en compte les variations saisonnières de fréquentation dans l'étude sur les petites lignes. C'est un ajout intéressant,

sur les lignes les moins fréquentées. Néanmoins, le rapport ne doit pas se limiter à cela, selon nous. Il devrait intégrer un volet portant sur le coût d'une remise à niveau des infrastructures et des préconisations pour permettre l'utilisation prolongée de ces lignes.

mais de la qualité de l'offre de transports et de la nécessité écologique. Tous nos citoyens sont dépendants du rail. Il faut par conséquent travailler à préserver toutes les lignes et à assurer un service de qualité. Il est d'ailleurs évident qu'une remise à niveau de ces lignes entraînerait une augmentation de leur fréquentation. En ne s'interrogeant pas sur ces deux points, le rapport demandé risque d'occulter la problématique du droit à la mobilité pour tous. Il nous semble donc indispensable qu'il aborde aborde la question de la mise à niveau des infrastructures et formule des propositions pour une exploitation prolongée des lignes du réseau secondaire, afin d'améliorer leur fréquentation. Quel est l'avis de la commission ? Le rapport

ne puisse être faite avant sa présentation. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Cet amendement vise à compléter l'étude sur les petites lignes par des préconisations pour chaque ligne. L'objectif de l'étude prévue à l'article 3 est de faire un diagnostic de la situation actuelle des lignes. Il paraît à la fois difficile et peu pertinent de définir des préconisations ligne par ligne dans le délai imparti, dès lors qu'il s'agit davantage d'un travail à mener par les pouvoirs publics à partir de ce rapport, notamment dans le cadre de la future génération de contrats de plan État-région, les CPER, s'agissant des investissements.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Vous avez dit, monsieur le sénateur Gay, que la réforme conduirait à l'abandon des petites lignes. Je veux redire, très solennellement et fermement, qu'il n'en est rien. Dès le départ, le Gouvernement a dit qu'il ne suivrait pas les préconisations du rapport Spinetta sur ce point. Ce sont bien

propose en faveur du ferroviaire. Il est prévu, au-delà de l'effort exceptionnel de 3,6 milliards d'euros par an,

un retard en 2017. Certaines lignes du réseau ferré font constamment l'objet de problèmes récurrents en termes de retards, d'annulations ou de ralentissements anormaux de parcours des trains. Selon un rapport de l'ARAFER de novembre 2017, en 2016, 11 % des trains des voyageurs sont arrivés en moyenne avec un retard d'au moins six minutes. Pour les voyageurs, cela représente 2 milliards de minutes perdues chaque année. Pour l'État, c'est une perte économique de 1,5 milliard d'euros d'euros par an. Afin d'identifier au mieux la source de ces problèmes, il conviendrait que le Parlement puisse disposer d'éléments susceptibles d'apporter des correctifs et d'informer utilement les usagers des lignes en question. Cet amendement vise donc à étendre la portée du rapport prévu à l'article 3 aux

de la commission ? Cet amendement vise à étendre le périmètre de l'étude aux lignes faisant l'objet de retards, de ralentissements de parcours et de suppressions de train récurrents. Il risque d'affaiblir la cohérence de l'étude demandée, en visant un périmètre excessivement large. Par ailleurs, je rappelle que les questions de qualité de service peuvent être traitées par les comités de suivi des dessertes.

qui correspondront au moindre mal, mais qui ne permettront pas d'assurer la qualité de l'égalité républicaine. C'est pourquoi nous préconisons qu'« en fonction des éléments du rapport, si une autorité propose la fermeture d'une de ces lignes, elle ne peut se faire qu'avec l'avis conforme du Parlement.

! Cet amendement vise à doter le Parlement d'un pouvoir d'avis conforme sur la fermeture d'une petite ligne, qui aurait été identifiée l'étude prévue à l'article 3. Rien que

de vote. Je n'avais pas compris que la réforme constitutionnelle prévue nous donnerait des pouvoirs aussi considérables J'avais plutôt le sentiment, madame la ministre, que le Gouvernement envisageait de les réduire quelque peu. Madame Lienemann, je partage votre passion républicaine. Or celle-ci tend à devenir, en tout cas dans cet amendement, totalement contradictoire. Vous voulez donner au Parlement

existent toujours et réunissent des élus autour d'une table, on a tout de même réussi à maintenir quasiment tous les points de contact de La Poste, que ce soit en banlieue ou dans le milieu rural. Si l'on avait délégué cette compétence au Parlement,

quant au sort réservé aux petites lignes- et dans les régions concernées, personne ne sourit ! -, l'article 3 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, une évaluation de l'état du réseau ferroviaire et des circulations sur les lignes les moins empruntées du réseau ferré national. du territoire et du développement durable a introduit dans l'étude proposée les critères d'« utilité collective » et de « contribution à l'aménagement du territoire », ce qui permet de ne pas limiter l'étude à une évaluation uniquement sous un angle financier et en termes de coût-avantage. Considérant que la préservation de ce patrimoine relève aussi d'un choix de société, les auteurs de l'amendement souhaitent disposer de plusieurs études et analyses afin d'éclairer de manière contradictoire et plurielle les enjeux concernant l'avenir de ces petites lignes, dans un contexte de forte évolution technologique, offrant de nouvelles opportunités. Des études socio-économiques devraient par ailleurs permettre une véritable appréciation des besoins en termes d'aménagement et de maillage du territoire, mais aussi de développement durable et de valorisation des externalités positives du rail par rapport au transport Pour toutes ces raisons, il est proposé de confier également au Haut Comité du système de transport ferroviaire et aux commissions parlementaires compétentes la réalisation d'études permettant de compléter l'évaluation produite par le Gouvernement.

Par ailleurs, il méconnaît le principe d'autonomie de chacune des assemblées parlementaires, car la loi n'a pas à définir le programme de travail des assemblées et de leurs commissions permanentes. L'avis est très défavorable.

Le projet de loi qui vous est soumis prévoit un rapport pour éclairer les décisions dans la perspective des prochains contrats de plan. Je ne suis pas certaine que nos concitoyens attendent de nous que l'on propose un deuxième rapport conduisant à des études dans les commissions de chacune des assemblées. Ils attendent de nous que l'on agisse, et c'est bien ce que le Gouvernement se propose de faire, plutôt que de multiplier les études et les rapports. Aussi, l'avis est défavorable.

: La parole est à M. Guillaume Arnell. Les conventions actuelles qui lient les opérateurs aux autorités organisatrices de transport sont très peu contraignantes sur les modalités de suspension des abonnements pendant les périodes perturbées et sur les dédommagements dus aux voyageurs qui ont été dans l'impossibilité d'utiliser l'offre de transport correspondant au coût de leurs abonnements. Il s'agit d'intégrer au code des transports la nécessité de prévoir, dans les conventions qui lient les opérateurs aux autorités organisatrices de transport, la possibilité, pour les voyageurs, de suspendre leurs abonnements en cas de grève ou de perturbations importantes et de prévoir la mise en place de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève ou de perturbation du trafic. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à imposer au sein des conventions de service public la définition de stipulations relatives aux droits des voyageurs en cas de grève. La généralisation imposée par l'amendement, en particulier pour la suspension des abonnements ou les dédommagements forfaitaires automatiques en cas de grève, mériterait de faire l'objet d'une évaluation de son impact pour les autorités organisatrices et leurs relations avec les entreprises ferroviaires.

Bien entendu, les critères de rentabilité et l'efficacité économique ont été mis en avant pour justifier le démantèlement de ce service public qui apportait, pourtant, beaucoup de satisfaction à ses usagers. Nous estimons qu'avant toute décision d'arrêt d'un tel service, particulièrement préjudiciable en période de congés, une mission parlementaire aurait pu se pencher sur la question.

Nous estimons qu'il faut redéployer les Intercités de nuit en desserte quotidienne pour recréer des liaisons ferroviaires qui ne passent pas par Paris, entre les régions périphériques. Cela permettrait, en outre, de désenclaver les zones de montagne ou encore les territoires excentrés. nous, une telle politique permettait d'encourager le report modal de l'avion sur le rail à l'échelle européenne, car les trains de nuit permettent de développer les liaisons ferroviaires internationales. Vous avez mis en avant la vétusté du matériel roulant. C'est malheureusement vrai. La SNCF a anticipé de longue date l'arrêt de ces trains, en ne réinvestissant pas. Mais nous touchons là à une question fondamentale des priorités données en matière de transports. Nous n'évoquons pas, par exemple, les investissements gigantesques en faveur de la route, qui sont contraires à une politique écologique cohérente et crédible. Ils sont d'autant moins évoqués qu'ils se font au profit du secteur privé, soit directement par la privatisation des autoroutes, soit indirectement en permettant aux transporteurs routiers de circuler avec une politique d'investissements minimum en infrastructures.

La suppression de ces trains pénalise les salariés qui, grâce aux trains de nuit, pouvaient préserver deux journées pleines de vacances. Quel

de diversifier l'offre de services de transports. Ainsi, si les services de trains de nuit répondent à un véritable besoin des voyageurs, des opérateurs pourront entrer sur le marché pour proposer de tels services. Il n'est donc pas utile de prévoir un rapport sur le redéploiement d'un service public de trains de nuit.

ils sont, en grande partie, le corollaire de la grande qualité de notre desserte TGV, qui a progressivement asséché le trafic des trains de nuit. Eh oui ! La SNCF n'a pas réussi dans le passé, et aujourd'hui non plus, dans le cadre de sa convention avec l'État à mettre en place un service de qualité ayant les faveurs de ses clients. Cela n'est pas, du reste, un problème propre à la SNCF puisque, vous vous en souvenez sans doute, le précédent gouvernement avait organisé un appel à manifestation d'intérêt qui n'avait pas permis d'identifier d'acteur alternatif intéressé. Pourtant, je veux le redire, l'État ne se désengagera pas des trains de nuit. Il continuera à soutenir les liaisons vers les régions qui ne disposent pas d'offre alternative. Aujourd'hui, ce n'est pas un rapport qui va résoudre les difficultés des trains de nuit, s'agissant en particulier de la qualité des sillons,

des rapports. En revanche, je veux dire ici très brièvement mon immense regret de la suppression, je le rappelle, de six trains de nuit- seuls deux ont survécu

Cet article prévoit la définition par ordonnance des modalités de l'ouverture à la concurrence en matière de tarifs, de conditions de vente et de gestion des gares. Il s'agit au fond de questions essentielles qui concernent la qualité du service aux usagers- vous le voyez, nous nous préoccupons également de ces derniers ! -et l'égalité d'accès au service public, dont la gestion des gares est un élément central. Toutes ces questions ne seront donc pas discutées au Parlement. Concernant les tarifs, et malgré la volonté de disposer de billetteries communes, de définir des tarifs maximums et de préserver les tarifs sociaux, nous craignons, au fond, comme cela s'est passé dans la majorité des situations d'ouverture à la concurrence de services publics, notamment dans le cadre de la téléphonie ou de l'énergie, que la multiplication des entreprises ferroviaires sur le réseau n'achève de déréguler les tarifs, qui, disons-le, sont déjà élevés et incompréhensibles. Nous avons d'ailleurs proposé des amendements à ce sujet. Nous notons avec inquiétude aussi le fait que les gares pourront demain être non seulement filialisées au sein d'une société anonyme, mais également gérées par des entreprises privées dans le cadre des contrats de service public passés avec les régions. une privatisation de lieux qui sont parfois, notamment dans des petites villes, de véritables centres de vie. Nous avons déjà largement parlé de cette question hier soir. Nous considérons que les gares font partie du patrimoine, des infrastructures, que leur gestion doit donc rester dans le giron de la SNCF et non pas être confiée à des opérateurs privés, qui n'ont aucune idée des contraintes d'exploitation de structures support service public. Nous voterons donc contre cet article qui enterre définitivement toute idée de service public dans le transport ferroviaire et qui, en organisant une nouvelle fois le passage par voie d'ordonnance, prive les parlementaires de leur pouvoir législatif. Vous comprendrez que cet exercice autoritaire du pouvoir, concernant l'avenir du service ferroviaire, nous semble inacceptable. La

qui traite des gares, pour partager ma passion et mon engagement sur ce sujet. Nous allons essentiellement traiter la question de la gare comme pôle d'échanges et de multimodalités, bref, comme centre d'organisation de l'intermodalité entre les transports. On peut aussi définir la gare plus largement, en allant au-delà du périmètre technique de la gare, comme un lieu de rencontre entre les deux cultures la culture du transport et la culture de la ville. C'est ce que l'on pourrait appeler la « grande gare ». Cette gare se caractérise par le fractionnement des acteurs : plusieurs autorités organisatrices, plusieurs propriétaires en gare, plusieurs exploitants. donc très compliqué d'organiser les gares. Nous nous limiterons, dans cet article, aux pôles d'échanges multimodaux, les PEM, c'est-à-dire à l'intermodalité. Mais nous pouvons nous intéresser plus largement au concept d'aménagement, et je fais le rêve, madame la ministre, que les projets soient tous centrés autour du voyageur.

Ces gares se caractérisent par des retards d'investissement, même si, au cours de la dernière décennie, ont émergé plutôt de beaux projets. Bref, ce sont des lieux

plaider en faveur d'une stratégie nationale pour ce qui pourrait être des nouveaux coeurs de ville. J'en suis convaincue, dans les petites villes et les villes moyennes, comme dans les villes de la périphérie parisienne, il existe un énorme potentiel pour

et d'harmoniser les contraintes d'exploitation des services de transport ferroviaire ainsi que les règles générales applicables à toutes les entreprises ferroviaires fixant des obligations de service public, notamment les tarifs sociaux, les règles en matière d'assistance ou d'indemnisation des voyageurs, le présent article met en relief les risques potentiels de dégradation de la qualité de service qui s'attachent à l'ouverture à la concurrence. Deuxièmement, cet article est également particulièrement dangereux sur la question des gares, en permettant aux autorités organisatrices d'intégrer la gestion des gares dans les contrats de service public. Nous ne souhaitons pas que les gares, outils d'aménagement du territoire et supports du service public, puissent être gérées ou exploitées par une entreprise privée, soumise à des impératifs de rentabilité financière.

Quel est l'avis de la commission ? Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? avec l'opposition à l'ouverture à la concurrence que vous avez manifestée depuis le début de ce débat. Je veux vous signaler qu'il s'agit d'une habilitation résiduelle puisque les principes de l'ouverture à la concurrence sont désormais inscrits dans le texte de loi lui-même, grâce aux concertations qui ont été menées et aux débats qui ont permis d'enrichir le texte. L'amendement est cohérent avec votre position. Je comprends Je comprends moins bien l'amendement du groupe socialiste, dont finalement je ne sais plus très bien s'il est favorable, ou non, à l'ouverture à la concurrence.

Nous proposons une rédaction très claire de l'alinéa 2 de l'article qui interprète un règlement européen de 2007 portant notamment sur les tarifs maximaux pour les voyageurs. Malgré les évolutions négatives de la tarification, l'État joue encore un rôle prépondérant en la matière au travers d'un encadrement des tarifs TGV et de l'obligation faite à la SNCF de pratiquer certaines tarifications sociales- nous les connaissons : famille nombreuse, congés annuels. Le rapport Spinetta préconise de mettre un terme à ces régulations administratives, tout comme il recommande d'augmenter la contribution de l'usager dans le coût du transport, un passage que tout le monde a bien lu ... Le rapport Duron est plus précis et et fixe à 50 % la part que devrait payer l'usager, ce qui représenterait par exemple une augmentation de 50 % à 100 % du prix du billet TER-Transilien. C'est tout de même une affaire sérieuse ... Dans un contexte de diminution drastique de la compensation de l'État à la SNCF pour les dépenses liées à la mise en place d'une tarification sociale sur les liaisons nationales, prévue dans le budget de l'État- la compensation est passée de 115 millions d'euros en 2004

les prescriptions tarifaires applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire ne manquent d'ambition. L'amendement que nous vous soumettons permettrait : le passage à deux enfants pour pouvoir bénéficier de la carte famille nombreuse qui permettrait 50 % de réduction

C'est bien pour cela que nous avons introduit à l'article 3 le principe d'un cadre législatif qui s'appliquera à toutes les entreprises ferroviaires, aussi bien au groupe public qu'aux autres opérateurs privés. Ces mesures visent précisément à garantir les bases d'une tarification sociale dans le cadre d'un marché qui sera prochainement ouvert à la concurrence. Monsieur le sénateur, votre préoccupation est, me semble-t-il, satisfaite. Je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Céline Brulin, dont le mandat de sénatrice de la Seine-Maritime commence aujourd'hui 1 juin, à zéro heure.

M. Joël Guerriau. Cet amendement détermine les conditions de distribution et de commercialisation des titres de transport dans le cadre du nouveau marché de transport ferroviaire de voyageurs. Il complète la rédaction de l'article 4, tel qu'issu des travaux de la commission du 23 mai dernier, en garantissant une concurrence libre et loyale aux entreprises de transport ferroviaire et aux distributeurs de titres de transport, en matière de distribution et de commercialisation des titres de transport. Il n'est en effet pas nécessaire que le distributeur soit une entreprise de transport ferroviaire pour que ces règles de libre concurrence s'appliquent à sa situation. Pour rappel, l'article 4 prévoit que les canaux de vente sont ouverts de manière régulée aux nouveaux opérateurs et vise à éviter que l'opérateur historique ne soit en mesure de privilégier ses filiales de distribution en matière d'information, d'accès aux billets ou de commissions, notamment par l'utilisation de sa marque ou de sa notoriété. Il est important de rappeler qu'en Allemagne les opérateurs alternatifs sont aujourd'hui confrontés à un opérateur unique qui contrôle l'accès à ses canaux de vente et impose, de fait,

Cet amendement vise à préciser que l'habilitation relative à la vente de titres de transport devra également assurer une concurrence libre et loyale entre distributeurs de billets. Il complète utilement la rédaction adoptée en commission visant les entreprises ferroviaires, notamment pour les distributeurs indépendants. L'avis est donc favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'amendement tend l'avis du Gouvernement ? L'amendement tend à préciser l'habilitation donnée au Gouvernement pour définir des règles en matière de distribution, en mentionnant le rôle joué par les distributeurs de titres de transport. Le texte actuel a pour objectif de mettre en place une concurrence libre et loyale entre les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, mais il ne porte pas sur l'ouverture à la concurrence de la distribution ferroviaire, marché qui est du reste déjà ouvert à la concurrence, avec en particulier de multiples agences de voyage physiques ou en ligne, et qui a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts de l'Autorité de la concurrence. Dans le cadre du marché de la distribution des titres de transport, il faudra porter une attention particulière au rôle des plateformes,

avec en outre la préoccupation de réfléchir à des tarifications multimodales, l'objectif étant de renforcer le rôle des régions dans ce domaine. Je vous propose,

Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Une gare est un lieu de vie, un élément de l'aménagement du territoire, un socle de l'infrastructure ferroviaire, qui doit rester sous maîtrise publique, ce qui n'est pas garanti si un opérateur privé devient titulaire du contrat de service public. La gestion des gares, nous l'affirmons, doit rester dans le périmètre de SNCF Réseau. Aussi, nous demandons que cette disposition soit exclue du champ d'habilitation de cette ordonnance.

De prime abord, cette habilitation peut sembler contradictoire avec l'article 1 A qui traite également de la gestion des gares. Ainsi, l'article 1 A permet de rassembler toutes les infrastructures, la voirie comme les gares, sous une unique responsabilité, celle de la société nationale SNCF. C'est une bonne chose. revanche, le pendant de cette réunification, c'est la filialisation de Gares & Connexions à laquelle nous sommes fermement opposés, car nous considérons qu'elle constitue un prélude à sa privatisation. Mais l'habilitation laisse entendre que cette gestion publique pourrait évoluer. Cette habilitation ouvre-t-elle la voie à la possibilité que d'autres exploitants puissent également gérer des gares ? Nous souhaiterions à ce sujet une réponse claire, notamment dans le cadre des contrats de service public, puisqu'ils sont évoqués. de cet amendement que l'on pourrait qualifier de précision, nous souhaitons donc apporter une garantie du maintien d'une gestion et d'une exploitation publiques des gares, ce qui semble somme toute assez logique si celles-ci sont exploitées par une filiale de SNCF Réseau

d'appel. L'amendement n° 115 vise à supprimer l'habilitation du Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les modalités de gestion et d'exploitation des gares. Or cette habilitation est utile, puisqu'elle doit notamment permettre aux autorités organisatrices de contractualiser directement avec les entreprises ferroviaires sur des objectifs en gare. Aussi, l'avis est défavorable.

que Gares & Connexions sera rattaché à SNCF Réseau, sous la forme d'une filiale. Cela garantit son caractère public, puisque son capital sera détenu par la société SNCF Réseau, qui sera elle-même intégralement détenue par l'État

gares permette de garantir un accueil optimal des voyageurs au sein des gares tout au long de l'année ou de favoriser la transformation des gares pour y permettre l'implantation d'autres activités en cas de fermeture. Je comprends parfaitement l'objectif de cet amendement, qui est de favoriser l'accueil en gare des voyageurs toute l'année, notamment en dehors des périodes de tourisme saisonnier. Toutefois, la rédaction proposée ne me paraît pas très claire et je doute de sa capacité à répondre aux attentes exprimées par les auteurs du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance qui fait l'objet de l'article doit permettre aux autorités organisatrices de contractualiser avec les entreprises ferroviaires sur des prestations en gare. Dans le cahier des charges de leur appel d'offres, les autorités organisatrices pourront donc fixer fixer des exigences sur les prestations à effectuer en gare, notamment en termes d'accueil des voyageurs ou de distribution des billets. Cela répond d'ailleurs en partie aux attentes des auteurs de l'amendement. Compte tenu de ces éléments,

L'amendement n° 117 vise à ce que le contrat de service public de transport assure le maintien des points de vente de billets dans toutes les gares du territoire national, ainsi que la présence d'un nombre d'agents suffisant. Vouloir que chaque gare dispose d'un point d'accueil physique et d'un agent pour assurer la vente de billets ne me paraît franchement pas réaliste, compte tenu de la diversité, en taille et en fréquentation, d'autant que, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, certaines entreprises ferroviaires pourront souhaiter proposer d'autres modalités de distribution des billets, par exemple la vente de billets directement dans les trains. La commission

réalisent, pour le compte de Gares & Connexions, des prestations en gare, comme cela est déjà possible aujourd'hui. C'est un facteur d'efficacité opérationnelle important

l'amendement n° 127 rectifié , les régions, en tant qu'autorités organisatrices des transports régionaux, décident du niveau de service qu'elles souhaitent. Il est important de leur laisser ce pouvoir de décision. Par ailleurs, les comités de concertation prévus pour les gares ou ensembles de gares permettront d'associer l'ensemble des acteurs, dont les collectivités locales et les usagers, aux politiques de services menées. Cette préoccupation me semble elle aussi satisfaite. Je sollicite donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai

Guillaume Arnell. Cet amendement prévoit la refonte de la procédure de fermeture administrative et de déclassement. Les éléments que doit contenir un dossier de fermeture ou de déclassement ont besoin d'être précisés à la fois pour sécuriser les décisions et pour ne pas créer d'incertitude juridique en cas de contestation contentieuse des fermetures : lien de la section avec le réseau, évaluation du potentiel de trafic fret et voyageurs réalisée par des experts indépendants, pertinence économique, sociale, énergétique, avis des comités de suivi des dessertes. Il est également prévu que ce dossier fasse l'objet d'une évaluation pour avis de l'ARAFER, autorité indépendante, avant l'avis conforme des régions concernées.

? Ces amendements visent à faire précéder les fermetures ou déclassements de lignes d'un dossier d'évaluation, soumis pour avis aux comités de suivi des dessertes, à l'ARAFER et aux régions concernées.

La procédure de fermeture d'une ligne est définie au niveau réglementaire et prévoit déjà la remise d'un dossier soumis à l'avis de la région concernée et des différentes parties prenantes. Par ailleurs, si le projet de fermeture se confirme, il est soumis à la validation du ministre des transports dès lors qu'il modifie la consistance du réseau ferré national. La procédure nous semble déjà suffisamment encadrée.

de variation des tarifs, notamment dans le commerce en ligne de transport, en fonction des heures de réservation. Depuis 1993, l'État a autorisé la SNCF à appliquer d'autres tarifications que celles qui sont liées à la distance kilométrique. C'est ainsi que les réservations TGV ont vu leur tarif modulé selon les créneaux

la CGT relève que ce procédé est peu utilisé chez les autres opérateurs européens et que l'on peut avoir jusqu'à cinquante tarifs différents à bord d'un même TGV

comme le révèle, qui a enquêté sur le sujet en février dernier. Avec la privatisation rampante, l'usage de ces méthodes se multipliera, toujours au détriment du porte-monnaie des usagers et toujours dans l'optique d'engranger un maximum de bénéfices dans un contexte de concurrence accélérée, alors que les incidences de la concurrence par les transports routiers, avec les fameux « cars Macron », se sont déjà exprimées. Dans ce contexte, il nous semble impératif d'abandonner la tarification de marché, pour revenir à une tarification au kilomètre. Quel est l'avis de la commission ?

Cette modification dépasse largement le périmètre du projet de loi, puisqu'elle s'appliquerait à toute vente de produits ou prestation de service en ligne. Par ailleurs, la pratique visée ne constitue pas, en soi, une pratique répréhensible. Enfin, le droit en vigueur comporte déjà des dispositions permettant, le cas échéant, de sanctionner des pratiques posant problème, notamment les pratiques commerciales déloyales. En conséquence, l'avis de la commission est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Madame la sénatrice, ? Madame la sénatrice, j'ai bien noté votre préoccupation, mais, comme vient de le dire M. le rapporteur, cette question dépasse largement le cadre de la réforme de notre système ferroviaire. Elle touche aux conditions de vente sur internet de manière générale. J'ai transmis au ministre chargé de l'économie votre souhait de voir évoluer le code de la consommation, mais je suis défavorable à votre amendement dans le cadre de la loi ferroviaire.

les pratiques commerciales trompeuses. Nous pensons qu'il est nécessaire de le compléter par une référence à la collecte de données personnelles en vue d'augmenter artificiellement les prix d'un service ou d'une prestation en ligne à l'occasion d'une connexion ultérieure. Cette méthode de marketing, communément appelée « », même s'il s'agit en fait de collecte de données plus larges que la seule adresse IP, a pour fonction de fournir des données sur le comportement d'un internaute sur une page web lors de sa visite sur un site

demande, mais l'incitation à effectuer un achat le plus rapidement possible, au risque de voir les prix continuer à s'envoler artificiellement. Nous considérons cette pratique comme

Quel est l'avis du Gouvernement ?

qui habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance les textes techniques du quatrième paquet ferroviaire, ces évolutions sont indispensables pour harmoniser les règles de sécurité ferroviaire dans le cadre de l'espace ferroviaire européen et faciliter l'arrivée de nouveaux entrants. L'avis de

parole est à M. Jean-François Longeot. L'objectif de cet amendement est de prévoir, dans le même temps que la transposition des directives européennes relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire et à la sécurité ferroviaire, la simplification de la réglementation en vigueur. En effet, ce travail de simplification réglementaire doit être mené parallèlement à un travail sur la simplification des référentiels de maintenance et d'exploitation aujourd'hui appliqués par SNCF Réseau. l'Association des régions de France a demandé au ministère des transports, dans un courrier daté du 5 avril 2018, la mise en place d'un groupe de travail portant sur la possible adaptation des référentiels de maintenance, afin d'engager une démarche de simplification réglementaire pour le transport de voyageurs sur les lignes locales. L'objectif final de ce travail de simplification est, vous le comprenez, une baisse des coûts de maintenance

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à ajouter un objectif de simplification aux mesures prises pour la transposition des directives techniques relevant du quatrième paquet ferroviaire. En commission, nous n'avons pas adopté cet amendement.

Il n'est pas certain que des modifications relevant de la loi soient nécessaires ; mais il ne faudrait pas que l'absence d'habilitation à procéder à des ajustements législatifs empêche des simplifications réglementaires qui en découleraient. Voilà pourquoi la

trop complexe. Or le chevauchement de nombreuses règles nuit non seulement au développement du transport ferroviaire, de voyageurs comme de marchandises, mais également à une bonne sécurité. À titre d'exemple, un conducteur qui devrait quitter le réseau ferré national pour rejoindre une voie de service portuaire pourrait être confronté à plusieurs régimes de sécurité rendant les normes à suivre peu lisibles.

? La commission a introduit cet article dans le présent texte pour autoriser expressément la création, par les acteurs du secteur ferroviaire, d'un groupement d'intérêt public, ou GIP, en vue de coordonner leurs actions destinées à renforcer la sécurité du système de transport ferroviaire. public exercera ses missions dans le respect des compétences de l'établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF Réseau : il n'a pas vocation à se substituer à l'État dans la définition des normes de sécurité applicables au réseau.

et tente de répondre à la problématique de la gestion de la sécurité liée à la multitude d'acteurs appelés à opérer sur le réseau ferré national. Créer un GIP ou plusieurs GIP pour coordonner l'action de ces acteurs en matière de sécurité, c'est reconnaître que l'ouverture à la concurrence pose problème. Si le statut d'un GIP est public, les acteurs privés peuvent en être partie prenante, voire y être majoritaires.

ont confirmé la nécessité d'une clarification du cadre social, non seulement pour les salariés qui pourraient être appelés à être transférés, mais également pour l'ensemble des salariés de la branche. Comme l'a très justement dit Mme la ministre en séance : « C'est un impératif non seulement d'équité, mais aussi de transparence, dans la perspective d'un arrêt du recrutement au statut. Dans ce contexte, la négociation collective entre les partenaires sociaux doit permettre de doter le secteur d'une convention collective qui garantisse un cadre social de très haut niveau pour l'ensemble des salariés. Cette négociation relève bien sûr de la responsabilité des partenaires sociaux. amendement vise à prévoir les mesures propres à favoriser la négociation collective au sein de la branche. Ces dispositions témoignent de l'importance des mobilisations, auxquelles

Négocie-t-on dans de bonnes conditions avec un pistolet sur la tempe ? Dans ce domaine, la manière forte me semble contre-productive. Ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas ?

et protecteurs pour l'ensemble des salariés de la branche. Ces malentendus étant levés, je vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai naturellement un avis défavorable.

cette précision dans la loi. Le code des transports prévoit d'ores et déjà de tels délais, par exemple pour l'avis rendu sur le document de référence du réseau ou dans les procédures de règlement des différends.

Cet amendement vise à rétablir des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et que la commission a supprimées afin de préserver le domaine de la loi.

liées à l'utilisation du réseau ferré national, en déterminant leurs modalités, les critères et la procédure de fixation, ainsi que les modalités de consultation de l'ARAFER sur ces questions.

qui ont une importance fondamentale en ce qui concerne l'utilisation du réseau, ainsi que le maintien ou non de l'utilisation de ce que l'on appelle couramment les petites lignes. En effet, si les modalités de détermination des redevances ne prennent pas en considération une volonté de maillage

Comme le souligne l'ARAFER, « la tarification des services conventionnés de voyageurs- TET, TER et Transilien -, qui relève d'une approche économique différente de celle des services non conventionnés, nécessite également d'être justifiée, pour des raisons qui ne sauraient exclusivement reposer sur l'objectif de conserver un même niveau de recettes à SNCF Réseau.

Depuis sa création, cette autorité a joué un rôle croissant et pris une place centrale dans le bon fonctionnement du système ferroviaire. En particulier, son avis conforme sur la tarification a été un aiguillon utile pour un régime de prix mieux assis sur les coûts et tenant mieux compte de la réalité des marchés ferroviaires.

En prévoyant de définir les modalités d'association et de consultation de l'ARAFER lors de la fixation des redevances, l'habilitation donnée au Gouvernement se révèle très large.

n'a vocation qu'à fixer le cadre applicable en matière de tarification, la détermination du niveau de redevance relevant de la compétence du gestionnaire d'infrastructure. Dans un souci d'équilibre entre, d'une part, le gestionnaire d'infrastructure, qui doit assurer le financement de ses coûts et, d'autre part, les entreprises ferroviaires, cet amendement tend également à permettre, en l'absence d'avis conforme de l'ARAFER, une reconduction des péages en vigueur, en leur appliquant au plus la hausse des prix à la consommation. en aucun cas d'un blanc-seing donné à SNCF Réseau pour contourner durablement un avis négatif de l'ARAFER. En effet, les tarifs applicables seraient au plus égaux

plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Ce serait autant de ressources en moins pour financer l'entretien d'un réseau dont vous connaissez les besoins.

Complétées en commission, ces habilitations permettront d'améliorer l'articulation de la fixation annuelle des redevances avec le contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau, dans un sens qui renforcera l'ARAFER. J'émets donc un avis défavorable n° 28 tend à supprimer le pouvoir d'avis conforme de l'ARAFER sur la tarification annuelle, ainsi que sa consultation sur le projet de budget annuel de SNCF Réseau. Ces restrictions affaibliraient significativement le rôle du régulateur. Or il est indispensable que l'ARAFER dispose de pouvoirs suffisants pour assurer une ouverture à la concurrence dans de bonnes conditions. Aussi, la

s'en tenir à ces modifications directes et précises au droit en vigueur, plutôt que d'apporter un ajout très général à une habilitation, lequel risque de ne pas se traduire par des évolutions concrètes.

souhaité donner, par ordonnance, un pouvoir d'avis conforme à l'ARAFER sur le volet tarifaire du contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau. Il s'agit là d'un point important, qui vise à assurer la cohérence du système tarifaire et à prévenir les difficultés d'articulation observées au titre de la tarification pour 2018. La rédaction adoptée n'exclut pas d'étendre cet avis conforme à d'autres éléments du contrat.

puissent être pris en considération par cette instance. En outre, aucun critère n'est défini à ce jour pour apprécier la soutenabilité d'une tarification par les entreprises ferroviaires : il est donc nécessaire de préciser ce point, notamment dans la perspective de l'ouverture à la concurrence. Aussi, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.

28 tend à supprimer l'avis conforme de l'ARAFER. Il me semble, au contraire, que cet avis conforme doit être maintenu. Le contrôle de la tarification par un organisme indépendant est une obligation fixée par le droit européen, et il s'agit d'un élément déterminant pour la réussite de la réforme que nous engageons. Le droit européen fixe un cadre clair de répartition des compétences des acteurs : l'État définit le cadre juridique de la tarification, SNCF Réseau élabore la tarification du réseau, et l'ARAFER la valide, en s'assurant que le montant et la structure des péages sont bien conformes aux règles applicables.

que les péages élevés pouvaient avoir sur le développement des trafics. L'intervention d'une autorité indépendante s'assurant de la soutenabilité des péages pour le transport ferroviaire est donc la garantie que les errements du passé ne se reproduiront plus : ce changement s'accomplira

Par ailleurs, alors que doit être visé un équilibre entre les redevances et le coût de gestion de l'infrastructure, je voudrais rappeler que les péages TER sont aujourd'hui très inférieurs à la quote-part du coût complet du SNCF Réseau qui leur est imputable, cet écart s'étant amplifié au cours des dernières années. Enfin l'adoption de l'amendement n° 136 rectifié modifiant l'article 1 garantit d'ores et déjà la prise en compte des spécificités des activités conventionnées dans l'évolution de la soutenabilité des redevances. Je suis donc défavorable aux amendements

afin que les décisions de cette autorité ne soient pas prises uniquement sous l'angle de la concurrence, mais puissent inclure, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, des considérations relatives à l'aménagement équilibré du territoire pour que ce collègue s'adapte aux problématiques actuelles. Le rail étant générateur d'externalités positives par rapport à la route, il paraît également opportun de « verdir » la composition de son collège en y intégrant un membre reconnu pour ses compétences en matière environnementale. Quel est l'avis de la commission ? Les effets de l'amendement ne sont pas clairs : s'agit-il de porter de sept à neuf le nombre de membres du collège ou de modifier sa composition à nombre stable ? Par ailleurs, la référence au domaine social et environnemental manque de précision. En tout état de cause, cette évolution ne nous semble pas nécessaire dès lors que les autorités compétentes pour nommer les membres du collège de l'ARAFER, notamment le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat,

Cet amendement vise à créer au sein de l'ARAFER un deuxième collège composé de représentants des élus du personnel des entreprises de transport ferroviaire, des usagers et des associations agréées de protection de l'environnement. En effet, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a fait évoluer la représentation des consommateurs et des usagers. Le présent projet de loi intègre cette évolution en soutenant, dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'amélioration de l'offre proposée aux voyageurs et aux chargeurs,

? Ces quatre amendements visent à doter l'ARAFER d'un second collège afin de représenter différents acteurs du secteur. Les amendements diffèrent par la composition de ce nouveau collège. Comme nous l'avons déjà dit en commission, le collège d'une autorité administrative indépendante comme l'ARAFER, dotée de pouvoirs que nous avons renforcés, n'est pas une instance de représentation du secteur mais un organe de décision pour assurer la régulation du secteur ferroviaire. Il est important de disposer d'un nombre réduit de membres exerçant leur fonction en toute indépendance. Le collège en toute indépendance. Le collège de l'ARAFER comprend actuellement sept membres dont la fonction est incompatible avec tout conflit d'intérêts dans le secteur ferroviaire. Créer un second collège constitué de représentants du secteur risque donc de compromettre le bon fonctionnement de l'ARAFER et l'indépendance de ses décisions,

Il est important que l'option ouverte au travers de cet amendement se limite bien aux lignes majoritairement financées par les régions, donc aux « petites lignes En effet, on s'aperçoit souvent que les prix estimés au départ dans le cadre des contrats de plan État-région peuvent doubler, ce qui fait effectivement augmenter la part financée par la région. Par ailleurs, le plus souvent la région avance

la ligne. Cet amendement vise à donner des outils supplémentaires à la région pour « challenger » le montant des travaux de SNCF Réseau et pour voir si une autre organisation avec les entreprises qui réalisent actuellement les travaux pour le compte de Réseau pourrait conduire à une baisse des coûts. tenu de l'importance des financements régionaux, il est légitime que les régions puissent choisir directement le prestataire en charge des travaux sans passer par SNCF Réseau. Quel est l'avis de la commission ? ? Cet amendement vise à permettre aux régions de demander à SNCF Réseau la délégation de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'entretien, de renouvellement ou de développement du réseau lorsqu'elles en assurent majoritairement le financement. L'objectif est de répondre à certaines situations dans lesquelles les régions sont en désaccord avec les coûts des travaux estimés par SNCF Réseau et souhaiteraient pouvoir elles-mêmes procéder à la maîtrise d'ouvrage- les régions nous font souvent Je partage la préoccupation des autorités organisatrices confrontées à ces difficultés qui conduisent parfois à hypothéquer l'avenir de certaines lignes. Lorsqu'elles financent la majorité,

Quel est l'avis du Gouvernement ? pour permettre la mise en oeuvre de modalités de gestion innovantes pour les lignes d'intérêt local et régional afin d'en réduire les coûts de maintenance et d'exploitation. On ne peut toutefois avoir une approche générique : dans certains cas la délégation de maîtrise d'ouvrage est appropriée, par exemple pour des travaux sur des lignes fermées avec peu d'interfaces avec l'exploitation du reste du reste du réseau, et dans d'autres elle l'est moins, par exemple, quand on a une forte imbrication avec l'exploitation ou encore avec d'autres projets. Je pense qu'il faut continuer le travail avec Régions de France

ans, la filiale de Vinci coûtera 250 millions d'euros par an à la SNCF, alors même que ladite entreprise a rompu son engagement de prendre à sa charge les 7,6 milliards d'euros de frais. Au final, c'est tout bénéfice pour cette filiale, qui n'a déboursé que 2,4 milliards d'euros et touchera encore 11 milliards d'euros sur l'ensemble de la concession. Chacun sait que les PPP représentent entre 10 et 20 % de surcoût

On supprime les rapports en commission et ils reviennent dans l'hémicycle ! Vous connaissez mon allergie

Nous estimons pour notre part nécessaire de maintenir le rapport du Gouvernement que prévoyait cet article afin de permettre au Parlement de disposer rapidement d'une évaluation du coût du remplacement du parc de locomotives au diesel fortement émettrices de CO2 par des motrices moins polluantes. Ce rapport pourrait constituer l'une des étapes importantes permettant de disposer d'éléments de diagnostic sur notre système ferroviaire, qui pourraient être mobilisés lors de prochains rendez-vous. Permettez-moi pour terminer d'attirer l'attention sur les petites lignes UIC 7 à 9. La plupart d'entre elles souffrent

l'avis du Gouvernement ? Je vous confirme que nous travaillons dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation sur les mobilités à un verdissement systématique des flottes,

d'expertise et de médiation destinée à explorer les solutions qui pourront être apportées sur la situation de ces lignes et les propositions qui pourront être avancées pour faire évoluer la réglementation à l'avenir.

Je n'ai pas bien compris la défense de l'amendement ...

et c'est normal : c'est la vie démocratique. Chacun a essayé de défendre son point de vue, avec ses convictions. Parfois on l'emporte, parfois on est battu. Il arrive aussi au rapporteur d'être battu

heures, débat sur le transport fluvial à la suite de la présentation du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du 1 février 2018.